La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 18 avril 2024 a été publié sur le site internet du Sénat.

et de sincérité du débat parlementaire. Dans quelles conditions démocratiques allons nous débattre cet après midi ? Les membres des commissions des finances des deux assemblées se sont vu communiquer une note confidentielle datée du 7 décembre 2023

Cette dissimulation, bien que préconisée par l’administration, est de nature à remettre en cause la sincérité du budget adopté à la fin de 2023 à coups de 49.3, sans vote par le Parlement. Le déficit est finalement de 5,5 % du PIB cette année. La procédure pour déficit excessif, que vous défendez par ailleurs à Bruxelles, pourrait donc s’appliquer à votre politique budgétaire. Excusez moi de le dire, messieurs les ministres, mais votre insincérité budgétaire se poursuit dans l’élaboration du programme de stabilité sur lequel nous allons débattre aujourd’hui. Ce document est censé retracer la politique du Gouvernement à court et moyen terme, et il doit être transmis à Bruxelles. Il est flou et insincère sur la forme : le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) doit contrôler les chiffres transmis a regretté que sa saisine ait été tardive, incomplète et qu’elle ne permette pas d’éclairer précisément les choix faits, alors que les finances publiques de la France sont dans une situation préoccupante. Ce document est flou et insincère sur le fond. Vous ne documentez rien,

Nous l’ignorons. Le programme des réformes, transmis en dernière minute, est un texte à trous, indigne d’un débat éclairé. L’insincérité de votre budget est vérifiable ; il nous en faut un nouveau. Un vrai débat démocratique s’impose,

je suis très heureux de vous retrouver pour présenter ce programme de stabilité, qui définit notre stratégie de rétablissement des finances publiques jusqu’en 2027.

Assez de cette manière systématique de peindre en noir la situation de l’économie française, des salariés, des industries et de tous ceux qui travaillent ! Je reconnais bien volontiers, monsieur le sénateur,

Il a fallu protéger, massivement et efficacement. Si c’était à refaire, je referais exactement la même chose.

ce serait irresponsable ! Si nous voulons que, demain, l’État puisse continuer à protéger en cas de crise, il faut mettre un terme aux dispositifs exceptionnels, relancer la croissance et réduire les dépenses publiques qui ne donnent pas les résultats attendus.

J’ai résisté à certaines demandes, et nous avons apporté les aides qui étaient indispensables. Merci ! Replongeons nous dans le contexte. À l’époque, Air France était menacée de faillite. Que fallait il faire ?

Les résultats sont là. Ah oui ! La France n’a pas connu de récession ; elle a amorti le choc inflationniste ; elle a été la première à retrouver son niveau d’activité d’avant la crise.

faut revenir sur le chemin du rétablissement des finances publiques, comme nous l’avions fait en 2017, 2018 et 2019. Tel est l’objet de ce programme de stabilité, qui est ambitieux puisqu’il doit nous amener à faire en trois ans ce que nous aurions dû faire en quatre : revenir sous les 3 % de déficit public en 2027.

de la croissance, des réformes de structure, de la réduction des dépenses là où cela est nécessaire parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Pourquoi est ce l’intérêt de la France

de considérer toute dépense de crise comme permanente, de confondre l’exceptionnel et l’ordinaire, dans une fuite en avant de la dépense publique dommageable à nos comptes et à notre nation.

pour les investissements indispensables dans la défense, dans la sécurité, dans la transition climatique, en évitant des dépenses moins utiles ou moins nécessaires. Le premier des réarmements doit être le réarmement financier.

Ensuite, le rétablissement des finances publiques entraîne deux conséquences positives majeures, que chacun doit bien comprendre. La première est le retour de la confiance des ménages et des entreprises,

des comptes publics bien tenus permettent d’obtenir une baisse des taux d’intérêt, qui allège la charge de la dette et soutient la consommation et l’investissement.

et des décisions à prendre, mais sur le cap à suivre, une fois encore, je tends la main à tous, car nous avons intérêt à nous rassembler. Enfin, moins de déficit et moins de dette, c’est évidemment moins d’argent pour les créanciers de l’État et plus pour les Français ; c’est éminemment souhaitable.

et de méthode. D’autres pays l’ont fait : la Finlande dans les années 1990, la Suède, le Danemark, l’Irlande, le Portugal plus récemment. Ce que tous les autres pays européens ont été capables de faire, pourquoi la France, au nom de je ne sais quelle mauvaise tradition historique, en serait elle incapable ? Il faut

à vous, avec Bruno Le Maire, à l’occasion de ce débat sur le programme de stabilité, qui actualise notre trajectoire macroéconomique et de finances publiques. Cette actualisation fait suite à un ralentissement de l’économie mondiale,

Malgré cette conjoncture moins favorable, les fondamentaux de notre croissance restent solides, soutenus par les réformes structurelles, les investissements mis en œuvre depuis 2017 et, de façon plus conjoncturelle, par l’accélération de la consommation des ménages permise par la baisse de l’inflation comme de leur taux d’épargne. Ce matin même, l’Insee a publié son estimation de croissance pour le premier trimestre 2024, qui est de 0,2 %, après 0,1 % au quatrième trimestre 2023. Notre acquis de croissance est donc de 0,5 % pour l’année 2024.

Pour atteindre cet objectif, nous réajustons notre trajectoire, avec une première marche crédible qui tient compte du double effet de l’exécution de 2023 et de la révision de la croissance pour 2024. L’objectif est de ramener le déficit de 5,5 % à 5,1 % en à 5,1 % en 2024. La suite de la trajectoire est également modifiée pour atteindre 2,9 % en 2027 : nous visons un déficit de 4,1 % en 2025, et de 3,6 % en 2026.

Ces économies ont été fixées en visant les dépenses publiques pilotables en cours d’année, mais aussi celles qui emportent le moins de conséquences sur notre croissance économique. Elles portent notamment sur l’aide publique au développement, sur MaPrimeRénov’ ou sur le compte personnel de formation. Nous avons également réduit les dépenses de fonctionnement de l’État et des opérateurs, pour un État plus sobre. Ces efforts nous ont déjà conduits à diminuer de 150 millions d’euros la facture énergétique de l’État, à céder pour 280 millions d’euros de biens immobiliers, et à diviser par trois les dépenses de conseil en deux ans.

Les ministères devront donc, sauf cas exceptionnel, exécuter leur budget dans le cadre des crédits disponibles, sans mobiliser cette réserve. Nous allons piloter la gestion au mois le mois, dépense par dépense, pour garantir

la même méthode. Ces mesures ne remettent pas en question les grands équilibres du budget pour 2024 : les dépenses vertes continueront à augmenter, et les budgets de la sécurité intérieure, des armées, de la justice, de l’éducation nationale et de la recherche progresseront encore. Concernant les collectivités territoriales, nous avons eu l’occasion, avec Bruno Le Maire, Christophe Béchu et Dominique Faure, d’affirmer une fois de plus devant le Haut Conseil des finances publiques locales (HCFPL), le 9 avril dernier, que la maîtrise de nos dépenses publiques restait un effort partagé. L’objectif pour les prochaines années, conformément à la loi de programmation des finances publiques (LPFP), entre 2024 et 2027, est que les dépenses de fonctionnement progressent un peu moins vite que l’inflation.

au même titre que la mission menée par le député Éric Woerth. Je demeure convaincu que c’est par le dialogue que l’État et les collectivités territoriales parviendront ensemble à construire des solutions face à la dégradation de nos finances publiques. Dans le champ social, nous poursuivrons nos efforts de maîtrise

les raffineurs de pétrole ou les laboratoires de biologie, des mesures seront prises en 2024, notamment sur la base des travaux des parlementaires, comme le Premier ministre l’a annoncé. Nous nous sommes d’ores et déjà engagés à travailler sur la question des énergéticiens et des rachats d’actions.

La croissance et l’emploi sont les meilleurs alliés de nos finances publiques. Malgré cette croissance solide, nous aurons encore un effort important à produire, prioritairement sur les dépenses, avec pour objectif de ramener le déficit à 4,1 % pour 2025. Pour y parvenir, nous devrons faire des économies dans tous les champs.

une fois encore devant la représentation nationale : dans la période que nous traversons et face à la conjoncture, cette nouvelle trajectoire reflète la détermination du Gouvernement à maîtriser la dépense publique, à tenir nos objectifs et à préparer l’avenir. La parole

présenté me paraît révélateur des errements et des renoncements du Gouvernement en matière de finances publiques. Revenons d’abord sur les performances économiques de notre pays. Certes, si l’on se limite à l’année 2023, nous faisons légèrement mieux que la zone euro,

l’économie italienne a crû l’an dernier au même rythme que la nôtre, et les économies portugaise, grecque et espagnole, par exemple, se montrent particulièrement dynamiques, avec une croissance comprise entre 2,3 % et 2,5 %, nous laissant loin derrière elles. Si l’on élargit

votre optimisme forcené ne saurait masquer le faible dynamisme de notre économie au regard de notre environnement immédiat et le scénario macroéconomique de ce programme de stabilité reflète encore ce biais.

En ligne avec ces hypothèses, vous évaluez la croissance potentielle à 1,35 % par an. Une nouvelle fois, ce scénario très optimiste n’est pas partagé par la plupart des conjoncturistes. Certes, messieurs les ministres,

–, vous vous réjouissez désormais des chiffres du premier semestre. Cependant, les faits sont têtus : le scénario macroéconomique que vous présentez est assurément trop fragile. Il ne me semble pas sérieux d’utiliser des prévisions non rigoureuses

En matière d’endettement public, les prévisions sont alarmantes : la dette, qui devait progressivement diminuer pour atteindre 108,1 % du PIB en 2027,

de l’année 2022, le Sénat avait adopté un projet de loi de programmation des finances publiques qui comportait un ajustement structurel inférieur et permettait pourtant d’atteindre une cible plus ambitieuse que

Au total, nous constatons combien l’effort à fournir est massif et sans précédent en un temps si court. Pourtant, comme l’écrit pudiquement le Haut Conseil des finances publiques, votre « documentation reste à ce stade lacunaire

que, même en prenant en compte le passage de l’Insee à la base 2020 au début de cette année, le déficit structurel est supérieur de plus de 0,5 point de PIB à ce qu’elle prévoit. À l’automne dernier, alors même que les prévisions pour 2023 étaient nettement meilleures que ne l’a finalement été l’exécution, je vous avais fait part des doutes de la commission des affaires sociales sur le volet de la LPFP En retenant les hypothèses de croissance du consensus des conjoncturistes, et en ne prenant en compte que les mesures effectivement documentées, la commission parvenait en 2027 à un excédent des administrations de sécurité sociale

Il est vrai que les programmes de stabilité sont, par nature, beaucoup moins précis que les LPFP. Par exemple, les dépenses et les recettes en points de PIB ne sont exprimées que pour l’ensemble des administrations publiques, et non par catégorie, ce qui constitue

d’autre part, il retient, surtout en fin de période, une hypothèse de croissance supérieure au consensus. Il n’est donc pas évident de savoir sur quoi nous débattons aujourd’hui. Faut il comprendre que le Gouvernement veut préserver la croissance, et donc ne pas faire d’économies aussi importantes ? Ou qu’il souhaite vraiment réaliser ces économies, ce qui réduirait immanquablement la croissance ? S’agit il pour nous de débattre de la nécessité de ramener le déficit sous le seuil des 3 % en 2027, du réalisme de cet objectif ou de la manière d’y parvenir ? Depuis un quart de siècle, les programmes de stabilité ont tous consisté en de simples projections, reposant sur des hypothèses conventionnelles, systématiquement optimistes. Nous pouvons donc discuter sans fin du réalisme de telle ou telle prévision, mais ce qui importe, en définitive,

Le Premier ministre a ainsi récemment annoncé une réduction de la durée d’indemnisation du chômage. Les déclarations publiques suggèrent en outre que le Gouvernement serait favorable à une diminution du coût des indemnités journalières et du transport sanitaire,

Ramener le déficit à 3 % du PIB en 2027 par des revues de dépenses dévoilées au fil de l’eau, sans jamais actionner le levier fiscal, semble irréalisable.

La vigie budgétaire indépendante chiffre cet effort à 2,2 points de PIB, soit environ 65 milliards d’euros. Si l’on prend en compte l’augmentation anticipée de la charge de la dette,

Gouvernement se voit placé, une fois de plus, à la merci des Républicains, qui agitent, tel un tigre de papier, le spectre d’une potentielle motion de censure sur le prochain texte budgétaire, que vous vous refusez à soumettre à la représentation nationale.

Si vous ne voulez pas écouter vos oppositions et votre propre majorité, écoutez au moins le Président de la République ! Au final, nous ne pouvons que nous demander qui pilote. Ça, c’est perfide ! Est ce le ministre Le Maire, qui veut imposer à ses propres partenaires politiques un collectif budgétaire avant les élections européennes ?

je le disais, plusieurs voix cohabitent, quand elles ne s’affrontent pas, au sommet de l’État. Il est vrai que cela finit par ressembler à une « foire à la saucisse », pour paraphraser celui qui en est le premier responsable.

Messieurs les ministres, les Français le sentent : le mur de la dette se rapproche et vous discutez de sa couleur. Pourtant, maîtriser nos finances publiques constitue une nécessité impérieuse pour faire face à la complexité des problématiques contemporaines qui se présentent à nous.

Ces investissements nécessiteront la mobilisation de moyens importants, que les leviers fiscaux actuels ne permettent pas de garantir. Nous devons faire le choix d’augmenter le niveau de solidarité pour financer les besoins sociaux, et de ne pas transférer l’intégralité du financement aux individus, au risque d’accroître encore les inégalités. Monsieur le ministre, la dépense publique ne saurait être considérée seulement comme un fardeau ; elle doit garder un sens redistributif, et continuer à assurer la gratuité d’accès à l’éducation et à la santé, tout en améliorant sa qualité. C’est fondamental pour contrer la montée du populisme. Sans une telle prise de conscience, vous condamnez notre pays au recul et vous poussez nos concitoyens vers les extrêmes. L’Histoire vous regarde et ne vous oubliera pas.

et je trouve que vous ne manquez pas d’aplomb. Vous êtes satisfaits de votre œuvre,… Il n’y a pas de quoi ! … pourtant, la situation budgétaire actuelle se caractérise par trois mots : le décrochage, la dissimulation, mais aussi la démission.

médaille d’argent pour les prélèvements obligatoires. C’est bien simple, notre pays ne brille désormais que par ses inconséquences. Quand on se compare, on se désole systématiquement. Sur l’endettement, seules la Grèce, qui se relève budgétairement, et l’Italie font désormais moins bien que nous. Emmanuel Macron aura même fait moins bien que ses prédécesseurs. Je me souviens

au niveau de l’Italie et de la Grèce. Nous sommes devant le mur : il vous faut trouver 95 milliards d’euros pour faire d’un déficit abyssal un déficit seulement catastrophique d’ici à l’alternance de 2027. Autant dire que la mission est impossible avec votre prisme idéologique.

ou limiter toujours plus la capacité d’investissement des collectivités, qui assurent pourtant 60 % de l’investissement public total et dont le rôle est central pour la transition écologique qui est sur toutes les lèvres

Vous préparez ainsi une cure d’austérité souterraine. Quand vous attaquerez vous enfin aux dépenses indues causées par l’immigration, par la fraude fiscale ou par la surcontribution au budget de l’Union européenne,

en matière d’économie, il y a deux excès à éviter : le premier, c’est l’excès d’optimisme ; le second, c’est l’excès de… L’excès d’optimisme consiste à considérer que tout va toujours pour le mieux, que l’avenir est radieux et qu’il le sera toujours. On y cède lorsque l’on se focalise sur les bonnes nouvelles et que l’on néglige les mauvaises. Il s’agit d’une forme d’irénisme qui peut se révéler coupable. On s’y complaît lorsque l’on manque de lucidité, lorsque l’on refuse de regarder un danger en face ou lorsque l’on ferme les yeux sur les causes de ce danger. L’excès de pessimisme est l’inverse : il consiste à tout voir sous un angle négatif, à tout critiquer par principe. C’est faire du mauvais temps une ligne de conduite. Ceux qui le pratiquent régulièrement ne savent plus comment réagir face à une bonne nouvelle : ils n’y voient même pas une éclaircie passagère, mais l’annonce d’une prochaine tempête, d’un désastre à venir. L’excès d’optimisme trahit une confiance aveugle en l’avenir, l’excès de pessimisme, une forme de défiance. Ces deux excès nuisent à la confiance, qui est la base de l’économie. Pas de commerce, pas d’investissements, pas de recrutement sans confiance en l’avenir. Or l’excès d’optimisme, comme l’excès de pessimisme, n’inspire pas confiance. Au contraire les responsables politiques qui s’y adonnent risquent le discrédit ; parce qu’ils font la part belle à l’idéologie plutôt qu’au pragmatisme, ils manquent en fait de lucidité. difficile de gagner la confiance lorsque l’on perd prise avec le réel. Vendredi dernier, les agences de notation Moody’s et Fitch ont finalement maintenu la note de la France. C’est une mauvaise nouvelle pour ceux qui se réjouissaient par avance à l’idée de fustiger de nouveau la politique du Gouvernement. Pour notre groupe, c’est une bonne nouvelle : une dégradation aurait pu alourdir la charge de la dette, qui est toujours la pire des dépenses publiques. mon sens, le sentiment qui devrait prédominer au Sénat. Je vous rassure : il ne s’agit pas de considérer les agences de notation comme les juges ultimes de nos politiques économiques ; en revanche, on peut raisonnablement considérer qu’elles ne cèdent ni à l’excès d’optimisme ni à l’excès de pessimisme. Elles ne notent pas l’état de nos finances publiques, qui résulte de décennies de laxisme budgétaire ; elles se prononcent non pas sur le passé, mais sur l’avenir. Vendredi, elles ont estimé que la France pourra rembourser sa dette. Pas plus, pas moins. Le programme de stabilité trace un chemin dans cette direction. Comme notre rapporteur général, je trouve que le rythme de réduction du déficit n’est pas assez rapide. Ce n’est pas exactement ce que j’ai dit ! En la matière, on va rarement plus vite que ce que l’on a annoncé ; souvent, on va plutôt plus lentement. Alors, autant faire preuve d’ambition ! Je crois tout de même que ce programme de stabilité ne pèche ni par excès d’optimisme ni par excès de pessimisme. Certes, la prévision de croissance est supérieure à ce que nous avons connu lors des dernières années, mais je note qu’elle est inférieure au rythme que connaissait notre pays en la matière entre 2017 et 2019, sous le gouvernement d’Édouard Philippe. Cette hypothèse de croissance, qui sous tend l’ensemble du programme, est donc réaliste. Bien entendu, elle dépend largement des événements géopolitiques, en Ukraine, au Proche Orient et particulièrement en Arménie – je reviens

L’important, selon nous, est de garder un cap clair : baisser les dépenses publiques pour réduire le déficit et amorcer le désendettement de la France. Notre groupe a fait plusieurs propositions en ce sens,

et nous avons un problème de crédibilité, que le Haut Conseil des finances publiques a illustré. Cela ne date pas d’aujourd’hui. Depuis vingt ans, il me semble qu’aucune loi de programmation des finances publiques n’a été respectée. Fort heureusement, les marchés achètent notre dette, qui reste un bon placement, mais cela ne pourra pas durer éternellement et la charge de la dette va devenir notre premier poste de dépenses. Nous avons un problème de crédibilité à propos de l’horizon des 3 % en 2027, qui paraît difficilement atteignable : nous n’avons jamais baissé la dépense publique de 0,5 point de PIB par an. an. Nous voyons mal comment assurer le réglage entre les coupes budgétaires, le soutien à la croissance, le maintien d’une trajectoire pro business, l’équité sociale et territoriale et la stabilité fiscale. C’est sans doute la quadrature du cercle. La recherche de ce bon réglage doit nous mobiliser, notamment pour ce qui concerne les coupes budgétaires nécessaires et le maintien d’un certain niveau de croissance.

car aller vers une crise politique qui s’ajouterait aux difficultés actuelles serait prendre un bien grand risque : les marchés financiers détestent ce genre d’incertitudes. Nous devons sans doute concentrer l’action des pouvoirs publics autour de quelques priorités, parmi lesquelles le redressement des finances publiques. nos concitoyens sont à juste titre inquiets quand ils mettent la somme des prélèvements fiscaux en regard de l’inefficacité de l’État sur bien trop de sujets. Le groupe Union Centriste reste une force de proposition, mais ne peut pas masquer ses graves inquiétudes.

nous débattons aujourd’hui du programme de stabilité qui présente les prévisions de croissance et la trajectoire des finances publiques que le Gouvernement s’est fixée à l’horizon 2027, conformément aux obligations du pacte de stabilité et de croissance de 1997. Rappelons le, ce pacte prévoit

pied. Dans ce contexte, que dire de la feuille de route du Gouvernement présentée dans ce programme de stabilité ? L’analyse économique du Haut Conseil des finances publiques, déjà abondamment citée, est sans appel : votre trajectoire pour nos finances publiques n’est ni crédible ni cohérente et vos prévisions sont si déraisonnablement

Pour réduire les déficits, vous disposez de deux leviers directs : baisser les dépenses ou augmenter les recettes. Depuis sept ans, vous décidez de priver le budget de l’État de milliards d’euros de recettes, en accordant des cadeaux fiscaux aux entreprises et aux plus aisés (ISF), exonérations de cotisations, niches fiscales, suppressions d’impôts et de taxes… De tels choix politiques emportent des dépenses fiscales considérables. Aussi, pour donner l’illusion d’une bonne gestion face à la Commission européenne et pour satisfaire les agences de notation, que vous chérissez particulièrement, vous n’actionnez qu’un unique levier : la réduction des dépenses publiques.

De plus, ce choix sacrifie le climat, la biodiversité et la lutte contre les dérèglements climatiques, dont les effets sont exacerbés par le fonctionnement néolibéral prédateur des grandes entreprises du CAC 40. Depuis sept ans, ces dernières voient leurs impôts et leurs cotisations fondre, pendant que les aides directes qu’elles reçoivent pleuvent, encore et toujours, sans contrepartie. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l’heure votre soutien à l’entreprise Renault. Comment votre gouvernement peut il s’en réjouir, alors que la nouvelle Twingo électrique, qui devait être produite

au programme de stabilité. De plus, le document que nous avons reçu est pour le moins lacunaire : vingt cinq pages, contre 247 l’an dernier, présentant un cap unique et inchangé : la « continuité des réformes réalisées depuis 2017

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, un gouvernement qui décide seul devrait assumer seul ! Cette décision solitaire s’est manifestée par la multiplication des 49.3 sur les projets de lois de finances et de loi de programmation des finances publiques. Les oppositions avaient raison : cette programmation était caduque avant même son adoption, elle est désormais dans un carton à Bercy ; toutes les projections macroéconomiques et les trajectoires de réduction de déficits qu’elle comportait ont volé en éclats. Décider seul, c’est aussi refuser de reconnaître que la politique de l’offre est une impasse. Les entreprises sont abreuvées d’argent public ; les dépenses de l’État ont progressé de 100 milliards d’euros depuis 2019 ; la croissance est atone ; les chiffres de l’emploi sont artificiellement gonflés par le million d’apprentis subventionnés ; la réindustrialisation serait à l’œuvre, mais la balance commerciale ne cesse de dévisser. Les entreprises se gavent de crédit d’impôt recherche,

La fin de la concurrence mondiale, la mise en place de barrières douanières européennes, de clauses de réciprocité, de protections, en somme, la fin du libre échange débridé, voilà les attentes des entreprises. Serons nous un jour « compétitifs », pour reprendre vos termes, face à la Chine ? Cela ne nous empêche pas d’être plus intelligents. 100 000 emplois devraient disparaître, avec la fin de la conjoncture post covid ; 68 000 défaillances d’entreprises sont attendues, alors que la marée des prêts garantis par l’État se retire. Le taux de chômage devrait s’établir à 8,4 % en fin d’année, alors qu’il est à 6 % dans l’Union européenne. La politique de l’offre n’ouvre décidément aucune perspective. Décider seul, c’est croire, enfin, que les finances publiques pourront se redresser sans améliorer les recettes publiques.

les 2,6 millions de salariés actionnaires perçoivent en moyenne un peu plus de 1 000 euros en dividendes par an. Ils ne seraient donc pas concernés. En revanche, selon France Stratégie, 0,78 % des Français raflent 94 % de l’ensemble des 63 milliards d’euros de dividendes distribués.

Vous voulez décider seul contre les oppositions, en feignant d’organiser des « dialogues de Bercy », des comités de concertation… Mais le débat parlementaire se tient ici, dans les hémicycles des assemblées, à visage découvert, là où chacun peut prendre ses responsabilités. Allons vers un projet de loi de finances rectificative et nous verrons qui propose quoi, qui vote quoi. Vous voulez éviter le débat avec les parlementaires ; vous avez si peur d’avoir raison avec nous que vous préférez avoir tort seul. Alors vous prévoyez, dans le programme de stabilité, des économies de 27 milliards d’euros en 2025, que vous n’avez pas étayées, qui sont d’une brutalité inouïe et dont personne ne veut, car la confiance est rompue. Nous ne vous en accordions guère, quant à nous, mais même votre partenaire s’impatiente. est bien que le ministre chargé des finances et le Président de la République débattent dans la presse, l’un préférant considérer le niveau des dépenses, l’autre les recettes en diminution.

se caractérise par l’incertitude des prévisions de croissance, par l’insécurité géopolitique et par la fragilité économique de nombreux ménages. Au fond, le principal problème de ce programme est qu’il n’a pas été écrit à partir de la réalité économique, mais à partir d’objectifs, ceux de Maastricht, vers lesquels nous entendons converger. Je ne me fais guère d’illusions sur l’utilité de ce débat non plus que sur sa capacité à infléchir les choix du Gouvernement. Néanmoins, je le crois important, car mon groupe politique est très attaché au projet européen, aussi perfectible soit il dans sa traduction concrète. Je le crois important, également, à un moment où l’état de nos finances publiques prend une dimension politique qui dépasse largement les seules controverses des économistes. Le coût exorbitant de la crise sanitaire, les révélations sur le déficit de 2023 – avec 21 milliards d’euros de recettes en moins –, les prévisions de croissance invraisemblables et finalement fausses, la dette publique en passe de devenir le premier poste de dépenses de l’État dans un tel contexte, l’inquiétude et le sentiment d’insécurité des Français ne sauraient être négligés. Ce que nous attendons du dialogue – sincère, pour le coup ! – que vous devriez avoir avec la représentation nationale, c’est la démonstration que l’orientation de nos finances publiques n’est pas un exercice comptable, mais bien un projet politique pour la Nation. Quel sens prendront la revue des dépenses ou la recherche de nouvelles recettes ? Bien sûr, le groupe RDSE se réjouit que la note de la France n’ait pas été dégradée par les agences Fitch et Moody’s. Force est de constater que la politique de soutien à l’activité a porté ses fruits et l’honnêteté intellectuelle, au vu des chiffres, commande de reconnaître que le chômage est au plus bas depuis quarante ans et que la réindustrialisation du pays a commencé. le projet politique que nous attendons désormais est celui du redressement et de la consolidation de notre modèle social et républicain, lequel est, ne l’oublions pas, un facteur majeur de notre résilience économique. Ce n’est pas moi qui le dis, mais des chefs d’entreprise de mon département. Ce modèle rassure les investisseurs et donne de la stabilité – c’est bien le mot ! – à notre économie. La crise sanitaire l’a d’ailleurs illustré. Cette consolidation pose évidemment la question des réformes et celle de l’efficacité de nos politiques publiques, car la dépense ne résout pas tout.

En résumé, messieurs les ministres, vous nous présentez un itinéraire : même cap, même destination, mais la pente promet d’être raide. Vous comptez sur une croissance du PIB supérieure à celle que projettent tous les prévisionnistes réunis. Cette ambition n’est pas hors d’atteinte, selon le Haut Conseil des finances publiques, mais elle est Vous misez sur le recul de l’inflation pour relancer la consommation des ménages. Je m’inquiète, pour ma part, du cap du million d’interventions pour impayés de factures d’électricité, franchi en 2023 : le médiateur national de l’énergie nous alerte sur le doublement de ses interventions pour ce Dans ces conditions, je ne suis pas certain que la confiance des ménages soit acquise. Par ailleurs, vous pariez sur la relance des investissements des entreprises, à l’heure où de nombreuses PME peinent à rembourser leur prêt garanti par l’État. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, au début du mois de janvier, votre ministère leur a permis de repousser leurs échéances, Reste, enfin, que les économies engagées par les annulations de crédits et le gel des réserves de précaution ne constituent pas une réforme structurelle, mais s’apparentent plutôt à un tour de vis dans le fonctionnement des ministères. Il s’agit d’une solution d’urgence et non d’avenir. La parole

ce début d’année 2024 nous a apporté son lot de mauvaises nouvelles économiques et budgétaires : une croissance pour 2023 légèrement plus faible que prévu – 0,9 % – et, surtout, un déficit budgétaire pour plus important que prévu – 5,5 % du PIB –, poussant notre dette à 110,6 % du PIB. Paradoxalement, cette dégradation du déficit public est en partie liée à une bonne nouvelle : le reflux de l’inflation. En effet, ce n’est pas un dérapage des dépenses publiques qui en est à l’origine, mais principalement une moindre rentrée de recettes fiscales, directement liée à une baisse de l’inflation plus forte qu’anticipée. Autrement dit, les cordons de la bourse sont tenus, mais les revenus sont trop dépendants d’aléas conjoncturels. Ainsi, les recettes des prélèvements obligatoires accusent une moins value de 21 milliards d’euros par rapport aux prévisions. Monsieur le ministre, l’objectif reste le même : le retour à un déficit budgétaire sous la barre des 3 % du PIB à l’horizon de 2027. Cependant, la tâche s’annonce ardue et les équilibres à maintenir, Dès février, constatant la dégradation des comptes publics, vous avez annoncé 10 milliards d’euros d’économies dans le budget de cette année et 20 milliards d’euros pour l’année prochaine. Le budget dédié aux outre mer comme les autres, mis à contribution à hauteur de 79 millions d’euros de crédits annulés. Pour autant, et je m’en félicite, il reste en forte hausse de 14 % sur un an avec 380 millions d’euros supplémentaires. Ces économies sont nécessaires pour éviter un dérapage plus important et montreront à nos partenaires européens, à la Commission européenne, aux marchés financiers et aux grandes agences de notation notre volonté de responsabilité budgétaire.

l’équilibre entre responsabilité budgétaire et soutien à la croissance sera au cœur de nos préoccupations dans les prochaines années. C’est pourquoi il me semble opportun d’œuvrer en parallèle, comme vous l’avez annoncé, à recouvrer les recettes fiscales escomptées initialement. Par exemple, la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, prévue pour rapporter 3 milliards d’euros en 2023, n’en a finalement rapporté que 300 millions. Monsieur le ministre, vous vous êtes exprimé sur le sujet et avez affirmé que le Gouvernement était prêt à améliorer le dispositif pour le rendre plus efficace dès cette année, à la hauteur des attentes. C’est une bonne chose. La hausse des prix de l’énergie ces deux dernières années, notamment de l’électricité, a fortement contribué à la dégradation de l’économie ; elle a eu un impact sur le pouvoir d’achat de nos compatriotes, sur la compétitivité de nos entreprises et,, sur le budget de l’État, en raison du coût des mécanismes de compensation et d’amortissement mis en place pour protéger les Français et les entreprises. Il est donc juste que ceux qui ont bénéficié de marges excessives au moment où les prix atteignaient des sommets participent au financement de ces compensations. Par ailleurs, la réforme du marché européen de l’électricité, en cours d’adoption, sans découpler complètement les prix de l’électricité et du gaz, devrait nous permettre de ne plus revivre à l’avenir ce genre de situation. Plus généralement, une meilleure évaluation de la dépense fiscale pourrait offrir des marges de manœuvre. Les outre mer ont déjà fait cet effort dans la loi de finances pour 2024 : certains dispositifs de défiscalisation les concernant ont été réévalués pour en améliorer l’efficacité et en diminuer les effets d’aubaine. Les revues de dépenses publiques prévues par la loi de finances pour 2024 devraient nous permettre d’effectuer une large remise à plat des dépenses budgétaires et fiscales de l’État. Les documents budgétaires affichent à ce titre une grande ambition, puisque ces procédures devraient permettre de dégager 6 milliards d’euros d’économies annuelles à partir de 2025.

s’agit évidemment d’une mauvaise nouvelle, mais celle ci doit s’apprécier au regard de notre situation et de cette ambition tout à la fois d’assainissement et de soutien aux investissements stratégiques, qui s’inscrit dans la logique des nouvelles règles budgétaires européennes, car notre économie peut supporter ce niveau de dette. D’ailleurs, nous pouvons constater que les agences de notation n’ont pas abaissé la note de la France. Les négociations à venir avec la Commission européenne et leurs conséquences Une procédure pour déficit excessif sera t elle ouverte ? Nous pouvons regretter que la réforme des règles budgétaires de l’Union européenne adoptée en début d’année ne permette pas de sortir les investissements pour la transition écologique du calcul de la dette.

La priorité doit aller à la croissance, à l’emploi et au pouvoir d’achat. C’est notamment ce qui a justifié la politique du « quoi qu’il en coûte » ou la mise en place du bouclier tarifaire énergétique. En la matière, la politique du Gouvernement est une réussite : le taux de chômage est au plus bas et le taux d’emploi n’a jamais été aussi élevé. Le signe le plus évident de cette situation est la disparition du chômage des principales préoccupations des Français. La politique conduite depuis 2017 porte ainsi ses fruits. La France est devenue la nation la plus attractive d’Europe pour les investissements étrangers, elle connaît une croissance positive, hors le trou d’air de 2021. Les créations d’entreprises sont au plus haut – 400 000 par an – et nous avons créé 2 millions d’emplois, dont 100 000 emplois industriels. Nous assistons au retour de l’industrie dans le paysage économique français, avec six cents usines ouvertes. Il ne faudrait pas qu’une politique budgétaire et fiscale trop restrictive vienne compromettre ces bons résultats. C’est en cela que la trajectoire présentée dans ce programme de stabilité est cohérente et réaliste. La parole

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le programme de stabilité budgétaire que nous examinons aujourd’hui intervient tout juste un mois après l’annonce du dérapage inédit du déficit public pour l’année 2023. Comme cela a été abondamment évoqué lors des interventions précédentes, ce programme a fait l’objet de vives critiques de la part du Haut Conseil des finances publiques. Non seulement la trajectoire budgétaire prévue n’est pas considérée comme crédible à court à court terme, mais elle s’avère surtout non soutenable à moyen terme et elle ne permettra pas de mobiliser les financements indispensables pour répondre aux enjeux de notre pays : la transition écologique et la réindustrialisation. En réalité, monsieur le ministre, tant que vous persisterez dans cette politique de désarmement fiscal, votre trajectoire budgétaire ne sera qu’un mirage qui abîmera encore davantage l’état de nos finances publiques.

Pourtant, vous persistez et vous signez : vous présentez une nouvelle trajectoire budgétaire envisagée sous le seul angle de la réduction des dépenses. Que nous dit la littérature économique à ce sujet ? Que la réduction de la dépense publique peut avoir un effet récessif. Selon l’OFCE, l’annulation de 10 milliards d’euros de crédits budgétaires cette année retirerait 0,2 point de PIB. Les 20 milliards d’euros prévus pour l’an prochain pourraient, eux, impacter la croissance de 0,6 point. Cela est d’autant plus préjudiciable que la bonne santé de nos recettes est étroitement liée à la croissance, socle fondamental du financement de notre modèle social. La « voie française » que vous dessinez est une impasse. Écoutez donc les économistes, les institutions qui suggèrent d’explorer de nouvelles pistes, comme l’OFCE, qui recommande une augmentation de la fiscalité, en veillant bien sûr à ne pas alourdir le fardeau pour les classes moyennes et les plus de nos concitoyens. Comment ne pas être convaincu de cette nécessité, quand le taux effectif d’impôt sur le revenu des trente sept ménages les plus aisés de France se limite à 0,26 % seulement, selon l’économiste Gabriel Zucman L’évidence est de retrouver des marges fiscales, de réintroduire un impôt sur la fortune, d’instaurer une taxe sur les rachats d’actions. Il est indispensable de mettre en place une véritable taxe sur les superprofits et de rééquilibrer enfin la fiscalité entre travail et capital. En ce qui concerne les dépenses, vous avez l’embarras du choix. Nous vous présentons quelques pistes : réduire les dépenses considérées comme antiécologiques, supprimer certains allégements fiscaux

portant sur un budget pour protéger les Français et préparer l’avenir. Comme d’habitude, les premières victimes de vos politiques budgétaires seront la transition écologique et les classes moyennes et, comme d’habitude, vous contribuerez à nourrir la défiance des Français à l’égard de l’impôt, de l’impôt, avec les risques démocratiques que cela comporte. Ce programme de stabilité porte en lui, en réalité, tous les risques : déstabilisation de l’économie, injustice sociale et renoncement aux ambitions environnementales. Il nous nous conduira certainement à de l’injustice sociale supplémentaire, sans doute à de l’instabilité budgétaire, et il ne nous empêchera pas d’être le cancre de la zone euro. La parole

La trajectoire de croissance est revue fortement à la baisse ; la prévision du déficit public est portée à 5,1 % du PIB en 2024, soit une augmentation de plus de 20 milliards d’euros par rapport à celle qui Comment ne pas s’étonner d’un tel réajustement ? Comment ne pas mettre en doute la crédibilité des prévisions du Gouvernement, voire leur sincérité, dès lors que celui ci semble avoir été informé dès le 7 décembre dernier que le déficit public pourrait s’élever à 5,2 % et non plus à 4,9 % ? Si la trajectoire est revue, les conjoncturistes ne partagent pas davantage ce scénario que les précédents. Ainsi, le Haut Conseil des finances publiques considère que la trajectoire retenue pour le PIB potentiel est surévaluée. Il y a donc, selon lui, « un risque important que l’évaluation soit révisée nettement plus à la baisse et donc que la part structurelle du déficit soit à la hausse Il estime par ailleurs que la France restera parmi les trois pays les plus endettés de la zone euro. L’ensemble de la stratégie d’amélioration des comptes publics défendue par le Gouvernement repose donc sur des hypothèses qui ne sont ni documentées ni partagées par la vingtaine d’instituts composant le. Le de retour – même de justesse – du déficit sous la barre des 3 % en 2027 relève – vous le savez, monsieur le ministre – de l’incantation, de la communication et de la méthode Coué. Le Haut Conseil considère, en effet, que l’atteinte de cet objectif « manque de crédibilité », car elle « supposerait un ajustement structurel massif » qui nécessiterait « un effort d’économies » qui n’a « jamais été réalisé par le passé » et « la mise en place d’une gouvernance rigoureuse », condition « qui n’est pas réunie aujourd’hui ». Je crois que tout est dit

Pourquoi nous alimenter en permanence de prévisions qui ont prouvé qu’elles n’étaient pas crédibles ? Pourquoi avoir fait adopter une loi de programmation des finances publiques et un budget dont nous avions souligné l’absence de crédibilité ? Pourquoi avoir refusé les économies – 7 milliards d’euros ! – et les recettes supplémentaires proposées par le Sénat ? Pourquoi, malgré la situation, le Gouvernement continue t il chaque semaine d’annoncer des mesures qui aggravent notre déficit public ? Pourquoi continuer à vouloir réduire les recettes de l’État ? Tout récemment encore, le Premier ministre a confirmé qu’une baisse d’impôts de 2 milliards d’euros serait appliquée en 2025 Pour mémoire, la suppression de la taxe d’habitation, celle de la contribution à l’audiovisuel public et la baisse de la CVAE coûtent déjà 35 milliards d’euros par an à l’État. Pourquoi ne jamais reconnaître vos erreurs ? Pourquoi ne pas vous attaquer réellement à la baisse des dépenses publiques ? Pourquoi faire semblant de croire qu’il s’agit d’un simple problème de recettes qui seraient conjoncturellement moins importantes que prévu ? Pourquoi vouloir faire peser sur les collectivités locales une partie des conséquences de cette situation, alors que celles ci n’en sont absolument pas responsables ? Pourquoi refuser que le Parlement soit saisi de ces questions essentielles ? Voilà, messieurs les ministres, quelques interrogations sur lesquelles nous aimerions obtenir des réponses ! La parole

Je commencerai par répondre au rapporteur général de la commission des finances sur les performances économiques 2017 2024. Je ne suis pas spécialement optimiste, j’essaie seulement d’être réaliste et de rendre à la France et aux Français ce qui leur appartient ce qui leur appartient : leur résultat économique. Il se trouve que la croissance cumulée de la France sur la période 2017 2023 est la plus forte parmi toutes les grandes nations européennes : la croissance cumulée de l’Allemagne de 2017 à 2023 est de 3,7

connu et respecté, qui fait référence, ne cesse de proclamer depuis des semaines et des semaines que la France fera 0,5 % de croissance en 2024. Il l’assène sur tous les plateaux, dans tous les journaux, sur tous les canaux de télévision.

risques, multiplie les normes, les règles et la complexité administrative. Il faut libérer la croissance européenne ; c’est ce que nous essayons de faire avec le Président de la République. Là est le vrai débat ; là est le vrai enjeu.

la confiance des entreprises et des ménages, qui, dès lors, libèrent leur épargne et investissent au lieu de garder de l’argent de côté. Monsieur Cozic, vous nous vous nous accablez sur le mur de la dette, mais vous ne me semblez pas proposer quoi que ce soit pour le faire tomber, sinon des dépenses nouvelles et de nouveaux impôts. Notre stratégie est différente : nous refusons les augmentations d’impôt et nous croyons à la croissance, aux réformes et aux réductions de dépenses.

; c’est vrai, mais cela remonte à quelques années, pour ne pas dire à quelques décennies. Le premier décrochage a eu lieu pendant la crise financière de 2008 2010, avec vingt six points de dette supplémentaires.

; soit, au contraire, pour la première fois depuis trois décennies, nous rétablissons les comptes, en estimant que les dépenses exceptionnelles doivent le rester, qu’il faut réduire les dépenses et relancer la croissance pour reconstituer des réserves qui nous serviront en cas de nouvelle crise. Tel est le choix politique fondamental qui se joue maintenant ! Vous aurez compris que le nôtre est fait : c’est de rétablir les comptes publics.

pour les masseurs kinésithérapeutes, pour les commerces de gros, pour les entreprises de voyage, pour les discothèques, pour les entreprises industrielles de services textiles, et pour d’autres

je propose que nous inventions, ensemble, ce nouveau chemin, celui d’une France capable de dépenser quand c’est nécessaire et d’économiser lorsque la situation s’est améliorée. Le covid 19 est derrière nous, l’inflation est derrière nous

Vous invitez à mobiliser des ressources pour investir : vous avez raison également, c’est pourquoi nous proposons de mettre en place l’union des marchés de capitaux, afin que nos entreprises puissent grandir. Rejoignez nous sur ce point aussi ; il me semble que nous avons suffisamment de points communs dans les choix stratégiques pour ne pas nous opposer sur des choix anecdotiques.

Oui, vous avez publié en septembre 2023 un document de planification nationale, qui offre une stratégie cohérente et une méthode générale indispensables face à ce défi.

sauf erreur de ma part, le Parlement n’a jamais été saisi d’un texte cohérent et ordonné sur la planification écologique, c’est à dire sur les objectifs et les mesures envisagées en matière d’atténuation préventive du changement climatique, sur l’adaptation inévitable de notre pays à celui ci, sur les énergies,

de projets d’arrêté, un plan sur ceci, un schéma national sur cela, une stratégie générale sur le reste…le tout avec, bien entendu, les sigles et acronymes technocratiques qui vous passionnent : Pnacc3, SNB, PPE, Écophyto, SNBC… Force sigles, certes, mais aucune vision d’ensemble présentée à la représentation nationale ! Efficacité sur le pilotage, ensuite : là encore, comme trop souvent avec ce gouvernement, les pilotes, co pilotes et presque pilotes se croisent et s’entrecroisent : le Premier ministre et le

comme vous le savez, par des demandes de contributions financières adressées aux collectivités sur des actions dont nous aurons à peine discuté et qui seront, en fait, sélectionnées à Paris. En matière de planification écologique comme dans d’autres domaines, nous parlons de décentralisation et de responsabilités partagées quand vous parlez de « déclinaison » et de « mise en œuvre » locales.

enfin saisi, comme dans une démocratie normale, d’un texte complet, cohérent et précis traitant des différents sujets de la planification écologique – atténuation, adaptation, énergie, modes de production, déchets, agriculture, biodiversité – et détaillant nos objectifs et les contraintes et incitations nouvelles que le Gouvernement juge nécessaire d’instaurer pour les mettre en œuvre ? Deuxièmement, quand le Parlement sera t il saisi d’une programmation financière claire et réaliste sur la planification écologique nécessaire à notre pays ? L’effort à accomplir est estimé à 100 milliards d’investissement chaque année pour les dix ans à venir. Combien mettra l’État, c’est à dire le contribuable ? Combien mettront nos entreprises, c’est à dire les consommateurs ? Combien mettront nos banques, c’est à dire nos épargnants ? Combien mettront nos collectivités locales, c’est à dire nous tous ? Ce débat sera douloureux, mais il est incontournable, et c’est au Parlement de statuer. Troisièmement, à court terme, comment allons nous financer, selon vous, les indemnités RGA, le rachat des biens touchés par le recul du trait

engagerez vous un vrai dialogue, une vraie négociation avec les collectivités locales sur un partage des objectifs, des priorités, des calendriers et des financements – bref, un dialogue moderne et normal dans une République décentralisée face à un enjeu national ? La parole

mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à vous remercier de l’organisation de ce débat. La planification écologique et les COP régionales étant des sujets importants pour le Gouvernement, il est toujours bon de pouvoir les évoquer devant la représentation nationale. Je vous demande de bien vouloir excuser le ministre Christophe Béchu, retenu à Turin par une réunion des ministres du G7 sur la transition écologique et énergétique. Notre pays a traversé récemment des épisodes climatiques extrêmes, qui manifestent plus que jamais la réalité et l’intensité du dérèglement climatique que nous traversons. Du Pas de Calais aux Alpes Maritimes, nos concitoyens et les élus locaux ont subi de plein fouet ses conséquences.

pour que nous puissions atteindre nos objectifs de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport au Cet engagement de baisse de nos émissions est fondamental pour préparer un avenir habitable, non pas pour les générations futures – nous n’en sommes plus là ! –, mais pour nous mêmes et pour nos enfants. La bonne nouvelle est que nous avons fait la moitié du chemin. Le défi qui se présente à nous maintenant est de diminuer autant nos émissions en sept ans qu’en trente trois ans. Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous rappeler l’origine de la démarche de planification écologique.

en lien très étroit avec le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, et avec l’appui du secrétariat général à la planification écologique. cette démarche inédite dans le monde nous pourrons identifier tous les leviers qui nous permettront, secteur par secteur, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre avec la bonne intensité. Les COP régionales sont tout simplement la déclinaison territoriale de la planification écologique. Elles doivent permettre de mettre en œuvre de manière effective, dans les territoires, les objectifs que nous nous sommes donnés nationalement et sur lesquels la France s’est engagée internationalement. Les COP régionales sont donc l’incarnation de la philosophie adoptée par le Gouvernement : une écologie proche des territoires, une écologie qui laisse aux acteurs du terrain la responsabilité d’identifier les leviers d’action et de s’organiser en conséquence – en somme, une écologie de cohérence. Les COP sont une nouvelle façon d’organiser collectivement la transition écologique dans les territoires. Elles visent à créer un cadre commun qui permette un dialogue articulé entre les niveaux nationaux, régionaux, départementaux, intercommunaux et municipaux. Leur but est de faire émerger des actions qui relèvent des compétences des collectivités territoriales, mais aussi de valoriser les actions déjà engagées, car nous savons que les collectivités sont extrêmement actives en faveur de la transition écologique. L’objectif est que le territoire s’empare de la planification écologique. Il s’agit, je le redis, d’un dispositif inédit : les COP, coanimées par le préfet de région et le président du conseil régional, permettent de faire discuter tous les échelons de nos collectivités et de les engager collectivement et localement. Nous en attendons trois points de sortie : d’abord, un alignement des parties prenantes sur les objectifs de la planification écologique à l’échelle de la région ; ensuite, un état des lieux partagé du territoire sur les dynamiques en cours et les programmes déjà engagés ; enfin, un plan d’action cohérent et pragmatique qui tienne compte des initiatives prises par l’ensemble des collectivités et qui complète les actions éventuellement déjà engagées. En outre, tous les sujets ne pouvant pas être parfaitement traités en une seule fois et en un an, la liste des sujets à évoquer lors de la prochaine COP et les modalités de suivi devront en émerger. J’ai évoqué le pourquoi et le comment ; permettez moi désormais de vous faire un état des lieux du calendrier. À l’heure actuelle, les COP ont été lancées dans toutes les régions, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, avec des calendriers qui respecteront notre objectif de disposer de feuilles de routes d’ici à l’été prochain, ou juste après. Je me félicite que le calendrier de lancement ait préservé des temps de concertation en amont de la réunion des COP pour s’assurer de la bonne prise en compte des spécificités de chaque territoire. Pour tenir ce calendrier, nous avons également déployé un accompagnement spécifique par les services de l’État, qui a pris plusieurs formes comme le recrutement de secrétaires généraux de COP dans chacune des régions concernées et la mise à disposition d’outils en support de la méthodologie.

Cette phase a permis à chaque territoire de disposer d’une vue concrète et structurée du type d’actions mises en œuvre ; on a ainsi embarqué les collectivités dans les COP en leur permettant d’exprimer leur point de vue, ou encore

ce jour, plus de 120 groupes de travail ont été mis en place dans toutes les régions, avec plus de 160 heures d’échanges. Ces débats ont été ouverts à tous les acteurs de la société civile, des professions agricoles aux associations de consommateurs, en passant par le personnel hospitalier, les associations de protection environnementale, les chambres consulaires ou encore les syndicats forestiers. se sont structurés autour des six thématiques de France Nation verte : mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer, mieux consommer, mieux produire et mieux préserver et valoriser nos écosystèmes. Dans certaines régions, des groupes de travail transverses complémentaires ont également été mis en place pour traiter, par exemple, de l’adaptation au changement climatique ou encore des enjeux d’emploi et de santé.

; ils sont le cadre idéal pour mettre en œuvre les ambitions fixées par les COP à l’échelle de chaque bassin de vie. Les CRTE ont vocation à devenir le cadre de travail de droit commun entre l’État et les collectivités, sous la forme d’un contrat chapeau qui rassemble les programmes d’appui territorialisés comme Villages d’avenir, Territoires d’industrie ou encore Petites Villes de demain. Je terminerai mon propos en rappelant, même si vous le savez déjà, que la mobilisation des collectivités est absolument essentielle à la réussite de la planification écologique. Nous allons

que nos réserves quant à la planification très verticale mise en place par votre gouvernement. Concernant les COP régionales, je dois avouer que les réunions organisées par le préfet de Saône et Loire et le sous préfet de Charolles ont eu le mérite d’informer

de plusieurs alertes sur les enjeux agricoles liés à cette démarche, dans sa dimension territoriale. En effet, il est essentiel de permettre à l’agriculture de prendre toute sa place dans l’atteinte des objectifs de décarbonation, de préservation de la biodiversité et de production d’énergies renouvelables. À titre d’exemple, le secteur de l’élevage, très présent dans mon département de Saône et Loire, a déjà contribué, du fait de la décapitalisation à l’œuvre depuis plusieurs années, à une réduction des émissions de gaz à effet de serre correspondant à la moitié de l’objectif fixé. Derrière ce qui pourrait sembler une bonne nouvelle se cache une vraie crainte. Chercher à décarboner le secteur de l’élevage par une réduction de la production sur notre territoire serait à coup sûr une grave erreur, car cela induirait une augmentation parallèle des importations de viandes.

La profession agricole mène actuellement un travail fin sur la gestion des troupeaux, l’alimentation des animaux, la diminution de la fertilisation azotée et la réduction des consommations d’énergie, qui est en mesure d’accélérer la voie de la décarbonation pour atteindre les objectifs de baisse d’émissions de gaz à effet de serre sans diminution du cheptel. Par ailleurs, l’entretien des prairies et des haies joue un rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité et les 13 millions d’hectares de prairies et parcours sur lesquels pâturent les bovins constituent des puits de carbone irremplaçables. L’élevage bovin français est non pas un problème, mais une solution pour l’environnement et le climat. Madame la ministre, la territorialisation de la planification écologique permettra t elle de relever ce défi ? La parole est à Mme la ministre

d’azote minéral entre 2020 et 2030 ; deuxièmement, la promotion de l’élevage durable, qui doit se faire en maintenant les effectifs bovins actuels, ceux ci ayant déjà beaucoup baissé ; troisièmement, la décarbonation des bâtiments et machines agricoles, par exemple les serres. ajoutent les leviers d’augmentation de la capacité des sols à capturer le carbone, que ce soit par le développement de haies, le maintien des prairies ou le déploiement de pratiques de stockage. il faut mentionner les leviers de préservation de la biodiversité et de la santé, à savoir essentiellement le développement de l’agriculture biologique et la réduction de l’usage de produits phytosanitaires.

Cédric Chevalier. Madame la ministre, je suis fier que ma région, le Grand Est, ait été la première à territorialiser la COP, avec son dispositif Grand Est Région Verte, dont l’objectif était d’impliquer l’ensemble des territoires et acteurs locaux dans la planification et l’accélération de la transition écologique. En contribution à ce vaste chantier, la collectivité a adopté une feuille de route ambitieuse proposant quarante cinq mesures d’adaptation au changement climatique. Par la suite, la région a voulu, en lien avec le secrétariat général à la planification écologique, demander des autodiagnostics aux collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, afin de repérer notamment les consommations actuelles et à venir de gaz à effet de serre ou encore les actions envisagées sur les ressources naturelles.

Je rappelle que, en novembre dernier, lors d’un débat sur le thème de la déclinaison territoriale de la planification écologique, j’interpellais déjà le ministre de la transition écologique sur la nécessité de simplifier les démarches pour les collectivités, notamment pour les candidatures au fonds vert.

Territorialiser la planification écologique est une très bonne idée sur le papier, mais les derniers signaux envoyés par le Gouvernement sur les questions écologiques n’invitent pas à l’optimisme.

Les régions s’inquiètent à juste titre de cette potentielle pénurie de moyens. Cela vient renforcer un sentiment d’incompréhension déjà très présent chez nos élus, un sentiment qui s’aggrave face à la mise en pratique de certaines politiques environnementales.

En effet, trois ans après le vote de la loi, nous sommes toujours en train d’affiner les modalités de calcul de l’artificialisation des sols, nous sommes toujours en train de défendre des projets d’envergure nationale et européenne, pour lesquels l’enveloppe foncière est souvent insuffisante, et nous sommes toujours en train de dénoncer des modalités de calcul de consommation foncière qui ne prennent en compte ni la taille des communes ni les projets territoriaux… Bref, il est vraiment temps de stabiliser les règles du jeu. Madame la ministre, je vous

la COP régionale va rallonger la concertation en Pays de la Loire ». Si la COP régionale des Pays de la Loire a d’ores et déjà décidé de retarder la concertation du grand public, c’est que les élus locaux ne sont pas venus aux ateliers du mois d’avril dernier, pourtant lancés par Christophe Béchu, qui jouait à domicile en lançant cette COP régionale voilà quelques semaines. donc un véritable problème. D’ailleurs, madame la ministre, je vous rejoins sur le fait que nous ne tiendrons pas nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation sans les territoires, sans les régions

Pour répondre à cette question, deux conditions essentielles me paraissent devoir être remplies. En premier lieu, la gouvernance des COP revenant conjointement aux préfets et aux présidents de région, il est impératif de rappeler la nécessité d’impliquer et d’associer tous les échelons de collectivités de veiller à la solidarité entre les territoires qui, pour la plupart, ont déjà établi des feuilles de route – je pense notamment aux PCAET et aux PAT. Nombreux sont les élus locaux qui déplorent la période de concertation accélérée.

Ces coupes contrastent avec les propos du Président de la République, qui, lors de l’élaboration du budget pour 2024, a affirmé que le virage écologique ne pouvait plus attendre, ainsi qu’avec le rapport Pisani Ferry chiffrant à 34 milliards d’euros annuels les besoins en financement public de la transition écologique.

en 2023. Oui, des mesures ont été prises. Je comprends que vous m’interrogiez sur ce sujet, mais quoi de plus légitime que d’avoir baissé la dépense de l’État en 2024

joué par les collectivités territoriales dans la planification écologique. Celle ci devait s’appliquer et s’ancrer dans les réalités du terrain. Sa réussite devait dépendre, en grande partie, de l’acceptabilité des mesures proposées. Il en était de même de l’identification des spécificités de chaque territoire territoire régional au regard des défis de décarbonation, de protection et de restauration de la biodiversité. Depuis, nos régions s’inquiètent du manque de perspective et de cohérence des messages envoyés par le Gouvernement sur les questions écologiques. Suppression du ministère de la transition énergétique, coupe budgétaire de plus de 2 milliards d’euros de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », dont 500 millions d’euros pour le seul fonds vert, qui est quasiment le seul soutien financier de la transition écologique des collectivités territoriales, déjà touchées par la diminution des fonds DETR et DSIL. une logique inverse aux attentes de nos territoires, lesquels espéraient, plutôt sereinement compte tenu des enjeux et défis climatiques actuels, que leur panoplie d’actions serait élargie, notamment sur la restauration de nos réseaux d’eau potable, dont les fuites occasionnent chaque année la perte de 1 milliard de mètres cubes d’eau, soit l’équivalent de la consommation de quelque 19 millions d’habitants. Que nenni donc, alors que la plupart des COP en sont à l’élaboration de leur diagnostic et à l’identification des thématiques sur lesquelles faire porter les efforts, notamment

qui est notre feuille de route nationale sur le sujet, fixe également un objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau de 1990. Cet objectif doit d’ailleurs être révisé par la nouvelle SNBC pour s’aligner sur l’objectif européen du:

elles ont un rôle essentiel à jouer dans ladite planification qui doit s’appliquer et s’ancrer dans les réalités propres à chaque territoire. Nous saluons en ce sens l’investissement et l’ensemble des travaux du secrétariat général à la planification écologique.

De plus, au regard des remontées de terrain qui seront faites, cela supposera dans de nombreux cas un fort investissement régional. Quels moyens seront alloués aux COP régionales pour traduire ces remontées de terrain ? Peut on envisager davantage de décentralisation sur certains sujets ? Enfin, madame la ministre, nous demandons qu’un bilan spécifique soit établi dans les territoires d’outre mer. La parole

ensuite, sur l’abandon du projet de loi de programmation sur l’énergie et le climat, définitivement enterré la semaine dernière, alors même qu’il s’agit d’une demande de nombreuses collectivités territoriales, convaincues que la souveraineté énergétique ne pourrait passer que par un effort de programmation, d’économies d’énergie et d’investissements dans les renouvelables ; enfin, sur les coups de rabot budgétaires non concertés. Il s’agit donc bien d’une injonction contradictoire pour les régions : toutes soulignent que les leviers identifiés par le secrétariat général à la planification écologique

Les COP régionales sont un outil limité aux collectivités. Sur le terrain, cela ne peut constituer un effet d’entraînement puisque les ménages, les acteurs socio économiques et les acteurs de la société civile en sont écartés. Madame la ministre, ma question est simple : les COP régionales sont elles toujours une priorité ? Le temps investi par les collectivités territoriales sera t il vain ?

Dans celle du 4 avril dernier, elle n’est plus que de 200 millions d’euros. Surtout, je lis un changement de philosophie : « Compte tenu du plan d’économies nationales, l’enveloppe qui sera dédiée à ces actions sera de 200 millions d’euros. Elle servira, selon les besoins remontés des territoires à l’issue des COP régionales, soit à renforcer

Très majoritairement, les élus locaux, dans toute leur diversité politique et territoriale, et les acteurs du monde économique en sont conscients. Aussi sont ils pleinement déterminés à agir sans relâche pour préserver nos territoires, nos écosystèmes et notre planète. Encore faut il qu’ils en aient les moyens.

trajectoire et notre ambition restent inédites avec une progression des dépenses en faveur de la transition écologique de 8 milliards d’euros. Nous avons pour objectif l’efficacité, afin que chaque euro dépensé donne des résultats pour l’environnement.

Faut il ajouter une énième couche ? Comment définir une place opportune pour les COP régionales ? Comment ne pas lasser les élus de ces partenariats changeants, sans fin et souvent sans bilan, alors qu’ils sont en train de s’engager pour définir une ligne d’investissements au travers de la DETR, de la DSIL et du fonds vert et que leur mandat arrive à échéance dans moins de deux ans

Comment pouvez vous garantir la réelle fonction intégratrice de la seconde génération de CRTE avec des moyens financiers et d’ingénierie nécessaires, sans accumulation d’obligations réglementaires ? Une approche transversale des différentes politiques publiques est nécessaire, mais trop de couacs demeurent.

Les choix retenus de covoiturage, de réticence au renforcement des dessertes par car et de lente croissance des dessertes par train semblent davantage liés à la volonté de respecter un cadre financier prédéfini qu’à un objectif de baisse des émissions

– certainement plus tôt que prévu – sur la biodiversité et nous divergeons encore sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter une contamination future de la nappe d’Alsace. Ici, au Sénat, nous craignons que les travaux prévus et déjà engagés ne servent qu’à retarder cette contamination, sans en réduire le risque. En actant cette situation, nous ne ferions que léguer le problème aux générations futures.

savons désormais que les modélisations réalisées dans le cadre des études diligentées ces dernières années sont caduques, que les cuvelages vont céder prochainement et que la mine sera rapidement noyée.

Madame la ministre, les COP régionales ont été mises en place pour planifier des politiques publiques. Planifier, c’est prévoir, mais c’est aussi anticiper. Aussi, je souhaiterais savoir quels moyens seront alloués au dossier Stocamine dans le cadre de la COP Grand Est et quand seront réalisées les études prenant en compte la rupture des cuvelages

de votre département. À son arrivée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu s’est saisi du dossier sans aucun. Il a veillé à la plus grande transparence sur les informations dont il disposait

le confinement ferait peser un risque inacceptable pour les personnels humains devant intervenir dans la mine. Le délai de confinement est de quarante deux mois, sans aléas de chantier. L’hypothèse d’un retrait partiel de certains fûts, compte tenu de délais incompressibles, aurait permis de ne déstocker qu’une quinzaine desdits fûts, ce qui aurait

le ministre a travaillé avec les élus locaux sur un plan de confinement permettant d’assurer la protection des générations futures dans le cadre de ce confinement et de poser dès à présent les bases nécessaires pour mettre en œuvre la réversibilité, c’est à dire le déstockage futur de la mine, voulue par les collectivités. La

des nouvelles COP régionales que vous avez mises en place. Les collectivités territoriales sont en première ligne pour la transition écologique et jouent un rôle essentiel dans la planification, qui doit s’ancrer dans les réalités du terrain. L’acceptabilité des mesures est primordiale et les COP régionales ne seront utiles que si elles aboutissent à une adaptation des objectifs nationaux au tissu local. Reste un sujet incontournable : le mur d’investissement qui se dresse devant les collectivités locales et les particuliers. Aujourd’hui, le financement de la planification écologique pose question. Des territoires ont calculé que, pour remplir les engagements de la stratégie nationale bas carbone à l’échelle locale, il faudrait multiplier par trente les financements de leur agglomération et par trois les engagements de l’État. Or les financements publics et privés, prévus à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d’euros, restent insuffisants au regard de l’ampleur de la transition à effectuer. Les récentes annonces de coupes dans le budget de l’État et de votre ministère mettent en cause la capacité du Gouvernement à financer une transition que les collectivités ne peuvent en aucun cas supporter seules. La lisibilité de l’action publique et la sécurisation des investissements nécessitent une programmation pluriannuelle des financements : c’est un outil essentiel pour les élus locaux. les élus locaux. Pouvez vous nous assurer que vous travaillez à une loi de programmation des financements accompagnant la planification écologique ?

une doctrine nationale dont les débats sur les objectifs et l’évolution sont occultés à l’échelon parlementaire et dont l’évaluation annuelle est jugée par la Cour des comptes, dans son rapport de mars dernier, comme impossible, les conditions n’étant pas réunies. Les objectifs régionaux sont réclamés, comme l’indique d’ailleurs le rapport d’information de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation de mars dernier. Le fait de guider l’action avec des tableaux Excel où le relief des écrans informatiques s’est rapidement heurté à la déclinaison opérationnelle, donc territoriale, sans oublier son volet budgétaire. Comme le souligne la Cour des comptes, la transition écologique devra mobiliser des ressources publiques et privées ; les ménages, les entreprises et les collectivités territoriales supporteront une part importante des dépenses. Face au cadencement désordonné de textes de loi relatifs à différents sujets – nous sommes

d’opposition ?… Il en est ainsi décidé. En application de l’article 8, alinéa 3, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes pour cette commission ont été publiées.

qui fut sénateur du Bas Rhin de 2014 à 2020 et secrétaire du Sénat. Je veux saluer aujourd’hui la mémoire d’un grand homme politique alsacien, engagé et profondément attaché à son territoire. Fervent défenseur du conseil unique d’Alsace, il avait soutenu ce projet avec passion en 2013, souhaitant que l’Alsace « prenne son destin en main ». C’était un élu de terrain. Comme beaucoup d’entre nous, il était entré en politique en devenant conseiller municipal, avant de devenir maire de Preuschdorf en 1989. Pendant vingt ans, il resta à la tête de sa commune. il entra au conseil général du Bas Rhin en 1992 et en devint le président en 2008, et ce jusqu’en 2015. Depuis 2021, il était conseiller régional de la région Grand Est.

Il fut également un membre assidu et actif de la délégation sénatoriale aux entreprises. Chacun garde le souvenir de cet homme pas très grand,

Le ministre des armées répétait alors que le problème de la masse de forces conventionnelles ne se posait pas pour nous, puisque nous disposions de la dissuasion nucléaire. Or voilà qu’au détour d’une interview le Président de la République tient le discours inverse,

La dissuasion, c’est l’assurance vie des Français ; c’est aussi le fruit de leurs impôts depuis soixante dix ans, depuis que le général de Gaulle a souhaité que la France acquière son indépendance stratégique.

Quelles sont les prochaines étapes envisagées par le Gouvernement après ce ballon d’essai ? Que compte t il dire à nos partenaires, et avec quels objectifs concrets ?

garanti une pleine compatibilité entre l’indépendance de la dissuasion française et la volonté de préserver en toutes circonstances la liberté d’action du Président de la République,

le président Chirac avait déjà fait le constat que la dissuasion française, par sa seule existence, était un élément incontournable de la sécurité du continent. Le président Mitterrand l’avait également énoncé. En clair, le Président de la République a rappelé que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne, ce qui n’a rien de nouveau. La dissuasion nucléaire française est pleinement souveraine. Le Président de la République est le seul à décider de sa mise en œuvre la décision ne sera partagée avec personne. Par sa dissuasion, la France contribue à la crédibilité de la défense de l’Europe. La parole

ces derniers jours, des groupes d’étudiants et de militants ont manifesté dans l’enceinte de Sciences Po ou aux abords de la Sorbonne, en soutien à la Palestine. Ces protestations ont entraîné des blocages, ainsi que plusieurs occupations de sites universitaires, avec le seul et unique objectif de contester, non de dialoguer. Un retour au calme était nécessaire, alors que les étudiants passent des examens dans quinze jours. Les cours ayant repris hier, je tiens à saluer l’engagement du Gouvernement, qui a permis aux élèves de reprendre le travail. travail. Si ce mouvement a pour le moment été circonscrit à quelques campus, il faut nous interroger sur les causes de ces manifestations, ainsi que sur la méthode employée par ces groupes, qui

d’argumenter, d’être en désaccord, de faire valoir ses idées et d’en débattre, et même – qui sait ? – de changer d’avis. Pas quand tout est bloqué ! Pour autant, il est inacceptable de voir des groupes minoritaires tenter de bâillonner et d’exclure de leurs réunions des personnes ayant des opinions différentes des leurs. Aidés de leurs soutiens politiques de La France insoumise, lesquels sont venus les saluer pour attiser les flammes de la haine et de l’intolérance, certains manifestants se sont permis de stigmatiser une partie des étudiants. Dans un pays qui a érigé la liberté d’expression en liberté fondamentale, ce n’est pas tolérable

La parole est à Mme Vanina Paoli Gagin, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Nous assistons avec consternation et inquiétude à des opérations de manipulation de la part de pseudo mouvements étudiants au sein de nos universités. En première ligne, Sciences Po et la Sorbonne, temples de la connaissance et du pluralisme des idées,… Ça, c’est fini ! … sont prises en otage par une minorité radicale. Cette mobilisation a pris des proportions dangereuses à Paris comme dans le reste de notre pays. Nous ne pouvons tolérer l’occupation de locaux universitaires ni l’instrumentalisation politique des étudiants, et encore moins la profération d’appels à la haine antisémite. Au fil des années, on a baissé la garde sur la défense du pacte républicain. Aujourd’hui, cette situation désastreuse a pris une tournure très politique,

Ces lieux devraient être consacrés à la confrontation des idées, au débat raisonné, à la transmission éclairée. Nous faisons face à une forme de négationnisme intellectuel – j’ose l’expression –, diamétralement opposé à l’esprit des Lumières.

et restons fermes ! Madame la ministre, que pouvons nous faire de plus pour que notre université renoue avec son universalité ? Bravo ! La parole

c’est non ! Les universités sont des lieux d’études. Leur mission est trop importante et trop précieuse pour que l’on piétine leur image et que l’on empêche leur bon fonctionnement, en tentant d’importer cette mobilisation des États Unis.

les « Beauvau » s’enchaînent. Après le Beauvau de la sécurité et le Beauvau des polices municipales, votre ministère lançait mardi dernier celui de la sécurité civile, afin de faire le bilan du modèle français et de donner des perspectives. parallèle, une intersyndicale représentant neuf organisations de sapeurs pompiers appelle à une mobilisation nationale le 16 mai prochain. Il ne fait aucun doute que cet appel sonne comme un avertissement : il faut des réponses concrètes et efficaces aux carences financières et humaines que l’on dans nos départements respectifs. Comme cela a été dit ces derniers temps, l’un des éléments ayant mis le feu aux poudres au sein de la profession est la publication du rapport commun de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile sur l’activité des sapeurs pompiers volontaires,

C’est pourquoi la profession, faisant preuve d’un sens aigu de l’intérêt général, fait part de son refus de toute application de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail aux sapeurs pompiers volontaires.

est solide, agile et résilient. Nous sommes tous ici très attachés à nos pompiers. Depuis de nombreuses années, ce modèle a fait la preuve de sa capacité à proposer des réponses rapides et adaptées à des sollicitations opérationnelles toujours croissantes. Toutefois, vous avez raison, il faut regarder la réalité en face et reconnaître

qui est malheureusement absent. Le 28 février dernier, en marge du salon de l’agriculture, le Président de la République a tenu à faire savoir à la profession agricole de ladite outre mer que cette dernière n’avait pas été oubliée

passe aussi par cette ferme outre mer. […] Au cœur de nos paysages, de nos territoires, avec des spécificités propres à chacun, il y a un projet à bâtir et des défis parfois plus importants ». Présente lors

affirme avec force l’impératif de souveraineté alimentaire et la dimension stratégique de notre agriculture, partout, sur tous nos territoires. Il vise trois objectifs, qu’il est important de rappeler ici. Le premier est d’assurer le renouvellement des générations, car, sans forces vives, il n’y a pas de souveraineté alimentaire. Nous devons être capables de former les nouvelles générations aux métiers de notre agriculture, pour produire davantage dans un contexte climatique

La parole est à Mme Céline Brulin, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen des dividendes faramineux, ExxonMobil annonce vouloir mettre fin à ses activités chimiques à Port Jérôme sur Seine, en Seine Maritime, et vendre sa raffinerie de Fos sur Mer, ainsi que des dépôts de carburant. 647 emplois directs sont en jeu, voire plusieurs milliers si l’on tient compte des entreprises sous traitantes et de l’ensemble du tissu économique touché. Les ressources des communes du bassin d’emploi et de l’agglomération Caux Seine seraient elles aussi considérablement affectées. Le Gouvernement et même le Président de la République doivent faire pression sur le groupe. Comment accepter que celui ci continue d’avoir accès aux marchés français et européen,

dans l’industrie automobile. L’abandonner ferait perdre un peu plus de souveraineté encore à la France. Cela mettrait notre pays à la merci de productions issues de gaz de schiste américains ou venues d’Asie, dans les conditions environnementales et sociales que l’on sait. Monsieur le ministre, à quand la souveraineté en actes ?

Monsieur le ministre, nous attendons plus que des regrets. Nous parlons d’activités stratégiques. Le Gouvernement, qui s’y refusait jusqu’à présent, semble examiner la possibilité de reprendre les activités stratégiques d’Atos. Pourquoi ne pas

116 parlementaires issus de 15 pays ont été ciblés par une cyberattaque parrainée par l’État chinois. J’ai appris officiellement hier que je faisais partie des 7 parlementaires français concernés, aux côtés de nos collègues sénateurs Isabelle Florennes

Les investigations du FBI ont formellement attribué ces cyberattaques au groupe de hackers APT31, associé au renseignement chinois. Ces hackers font nommément l’objet d’un acte d’accusation du ministère de la justice américain depuis le 25 mars dernier. mars dernier. Il s’agit clairement d’un acte de cyberguerre, commis par une dictature 2.0. À moins d’une semaine de la venue en France du président Xi Jinping, nous sommes confrontés à une manifeste ingérence étrangère d’envergure de la part de la Chine,

vous formellement ces attaques à ce groupe, comme l’ont fait d’autres pays, et demanderez vous l’ouverture d’une enquête ? Prévoyez vous de renforcer l’assistance aux parlementaires, pour les protéger des États qui ne tolèrent pas la liberté d’expression et qui les menacent ouvertement ?

dans le cadre approprié nos préoccupations concernant les cyberattaques qui visent nos intérêts. Ces dernières font l’objet d’investigations au plan national, y compris d’un point de vue judiciaire. le Gouvernement n’exclut pas d’attribuer publiquement ces cyberattaques à un groupe donné, vous comprendrez que nous ne puissions pas, à ce stade, communiquer davantage sur ce sujet. Plus généralement, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour contrer ces menaces.

et Territoires. La semaine prochaine, le Président de la République recevra le président chinois, Xi Jinping. Je fais l’impasse sur la balade bucolique dans les Hautes Pyrénées sur le chemin des souvenirs d’enfance d’Emmanuel Macron,

qui concerne notre sécurité, l’espionnage chinois – c’est à dire une ingérence étrangère – s’invite dans notre hémicycle et dans la campagne des élections européennes, ce qui constitue une menace réelle pour la souveraineté et l’intégrité de l’Europe. Est ce au programme des discussions ? Enfin, les atrocités commises contre les Ouïghours exigent une action immédiate de la part de la communauté internationale. Le peuple ouïghour continue, au vu et au su du monde entier, de subir la répression et l’exploitation.

commet le gouvernement chinois sur son peuple. Nous devons accroître la pression sur la Chine pour mettre fin à ces violations, pour garantir l’accès à des observateurs indépendants et pour poursuivre les responsables. Comment le va t il, lors de cette visite du président chinois, réaffirmer les grandes valeurs de la France et son engagement envers les droits humains, la protection de notre démocratie et les droits fondamentaux des Ouïghours ?

Madame la sénatrice Guhl, vous évoquez la visite d’État du président Xi Jinping en France les 6 et 7 mai

les défis mondiaux, les enjeux globaux, les irritants commerciaux et la protection des droits de l’homme.

la biodiversité et de financement du développement. Sur les sujets difficiles, nous assumons d’entretenir un dialogue politique exigeant avec la Chine. Nous exprimerons clairement le caractère insoutenable du déficit commercial bilatéral et notre détermination à défendre nos industries et nos emplois. Par ailleurs, nous aborderons la situation des droits de l’homme en Chine.

de participer à la restructuration de la dette et d’apporter son conseil. Un mandataire a été nommé ; je l’ai reçu. Dès que les difficultés de ce groupe, qui compte 10 000 salariés et exerce des activités stratégiques, se sont renforcées,

j’ai déposé une offre d’intention pour acheter l’intégralité des activités stratégiques d’Atos et éviter que la moindre d’entre elles, que ce soit dans les supercalculateurs, dans la cybersécurité ou dans les transmissions sécurisées, notamment pour la défense, ne puisse passer

ce n’est pas parce que nous faisons les choses discrètement que nous ne les faisons pas efficacement. Ce n’est pas parce que nous travaillons dans le silence que nous ne prenons pas nos responsabilités. Il vaut mieux traiter certaines affaires discrètement, pour prendre les décisions au bon moment, comme nous l’avons fait. Monsieur le ministre, c’est bien tard et c’est beaucoup trop peu ! Vous ne pouvez pas nous parler d’intérêt vital et de souveraineté et regarder passer les trains depuis le début des difficultés du groupe.

Nous regrettons que l’hypothèse du maintien du groupe dans son entier ne soit presque jamais envisagée par les services de l’État et nous considérons que la solution proposée par le Gouvernement ne réglera pas la question de la soutenabilité de la dette et de l’avenir du groupe. Il nous apparaît indispensable d’éviter une procédure de sauvegarde qui signerait le début d’une vente à la découpe de l’entreprise et entraînerait un pillage de technologies stratégiques essentielles à notre souveraineté, alors qu’il est nécessaire de maintenir nos capacités de recherche et développement.

Nous sommes d’avis que l’État doit garantir l’ensemble des contrats publics du groupe Atos, afin de ne pas pénaliser encore davantage son activité. Enfin, nous demandons que l’État s’engage, au nom de la souveraineté, à renforcer le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France par le biais de sociétés, de fonds et de banques, en envisageant de restreindre, voire d’interdire, la vente à découvert sur les entreprises cotées ayant des activités souveraines. La parole

Quand la SNCF vous annonce, pour justifier un retard ou une annulation, l’absence d’agent d’astreinte, un vent trop fort, la présence de givre, de sangliers ou de feuilles sur les voies, vous n’êtes plus vraiment surpris par ces situations qui frôlent l’absurde. La réalité, monsieur le ministre, c’est que nos Intercités, ces trains du quotidien qui ont longtemps incarné l’aménagement équilibré du territoire, sont malades. Ils souffrent d’un sous investissement chronique depuis plusieurs décennies. La colère gronde sur toute la ligne, et nos territoires risquent de dérailler. Face aux galères de la SNCF et à défaut de pouvoir prendre le train, plusieurs de nos entreprises locales ont menacé de prendre le large. Dans ce contexte dégradé, les travaux de régénération et la mise en circulation des nouvelles rames Oxygène auraient pu redonner une bouffée d’air au matériel roulant à bout de souffle des lignes Paris Orléans Limoges Toulouse (Polt) et Paris Clermont Ferrand. Or la nouvelle est tombée en fin de semaine dernière : le constructeur nous informe d’une défaillance technique qui qui reporte la livraison au premier trimestre 2027. Ce matériel nous a initialement été promis pour 2022. Avez vous la garantie que ce nouveau délai sera respecté ? Toute la transparence doit être réalisée sur la responsabilité de chacun. Pourquoi avoir choisi un constructeur qui n’a pas l’habitude de travailler avec la SNCF et qui proposait un matériel sur plan, dont aucune des composantes n’avait été éprouvée ? Le sort s’acharne sur nous, puisque la SNCF envisage, semble t il, de suspendre le trafic de jour sur la ligne Polt entre Paris et Orléans d’août 2025 à janvier 2026 : confirmez vous ce scénario inacceptable ? Enfin, le Gouvernement a t il prévu de replacer ce dossier en haut de la pile pour sauver nos trains d’équilibre du territoire et promouvoir le moyen de transport le plus décarboné qui existe à ce jour ? Comment leur redonnerez vous la fiabilité, la rapidité et l’intérêt qu’ils méritent ? Monsieur le ministre, combien de temps encore allez vous nous laisser sur le bord du quai ?

Samedi dernier, la mort à Châteauroux de Matisse, 15 ans, poignardé par un autre mineur qui était déjà poursuivi pour des actes de violences avec armes, a montré l’incapacité de la justice pénale à répondre à l’ultraviolence chez les plus jeunes. Toutes mes pensées, auxquelles j’associe Nadine Bellurot, sénatrice de l’Indre, vont à la famille du jeune Matisse, à ses amis, ainsi qu’aux habitants et aux élus de Châteauroux qui ont été touchés par ce nouveau drame. Celui ci s’ajoute à une liste déjà bien trop longue de meurtres avec violence commis ces dernières semaines par des mineurs. L’enquête est en cours, la justice fait son travail, d’ores et déjà que les juges ne disposaient pas de moyens suffisants pour prévenir une récidive rapprochée et engager la responsabilité éducative des parents. des parents. Le code de la justice pénale des mineurs ne permettait pas aux magistrats d’apporter une réponse rapide et efficace pour éviter ce nouveau drame. Aussi, madame la ministre, qu’entend faire le Gouvernement pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise ?

un texte sur la justice pénale des mineurs est en cours de préparation et traitera de la responsabilité parentale et de la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs.

Face à tout cela, oui, nous devons continuer de travailler ensemble. Des concertations sont ouvertes, et le Premier ministre et tous les ministres concernés y prennent toute leur part. Je sais pouvoir également compter sur votre démarche et votre action en ce sens.

voyons toujours rien venir. Plusieurs fois inscrit à l’ordre du jour, l’examen de ce texte a été reporté. Le Sénat a pris toute sa part de responsabilité en formulant des propositions dès 2022, et la commission des lois engagera bientôt une réflexion sur l’exécution des peines, à commencer par les courtes peines. pour prévenir la violence, seule une réponse pénale ferme et rapide, exécutée dans des conditions adaptées aux mineurs, limitera la récurrence de l’horreur que nous avons connue à Châteauroux. Aussi, agissez, et le Sénat sera au rendez vous

le groupe Union Centriste. Ma question s’adressait à M. le ministre délégué chargé de la santé. J’y associe Jocelyne Guidez et de nombreux autres collègues de tous les territoires. La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), en coordination avec l’ensemble des syndicats de médecins libéraux, annonce une grève totale à compter du 3 juin prochain.

La parole est à Mme la ministre déléguée chargée du renouveau démocratique, porte parole du Gouvernement. Madame la sénatrice, vous interrogez le Gouvernement sur l’avenir de l’hôpital privé dans le contexte des réactions du secteur privé aux annonces des tarifs hospitaliers pour l’année 2024. Les établissements de santé privés ont bien évidemment toute leur place dans l’offre, pour répondre aux besoins des patients et des Français. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d’une campagne tarifaire équilibrée, qui repose sur les mêmes principes et sur les mêmes paramètres pour tous. La prolongation du mécanisme de sécurisation des recettes s’appliquera au secteur public comme au secteur privé. Certaines activités, comme les maternités, bénéficieront d’une revalorisation plus importante de leurs tarifs, dans le public comme dans le privé.

et de la recherche. Madame la ministre, Sciences Po n’en finit plus de sombrer dans une dérive idéologique, très loin de l’idéal de son fondateur, qui voulait en faire un lieu d’excellence et d’accès au « culte des choses élevées », comme il disait. Depuis les attentats du 7 octobre, on ne compte plus les incidents, les conférences annulées et les blocages de site. On a même assisté à l’exclusion d’une étudiante juive, préfiguration d’une nouvelle forme d’apartheid dans le microcosme de la rue Saint Guillaume. Vendredi dernier, après l’occupation du site de Paris, la direction a failli. Elle a cédé face à 200 agitateurs convaincus d’être dans le camp du bien, mais nullement représentatifs des quelque 15 000 étudiants de l’institution. Elle a abdiqué devant une poignée de jeunes qui n’hésitent pas à afficher leur soutien aux terroristes du Hamas et qui brandissent leurs mains rouges en hommage aux bourreaux des soldats israéliens de Ramallah. Elle s’est soumise, enfin, au diktat d’un comité d’ultragauche, dont elle a d’ailleurs repris le verbatim importé des

C’est pourquoi des campus sont évacués lorsqu’ils sont bloqués. Je voudrais citer l’évacuation de la Sorbonne hier, celle du campus Saint Thomas de Sciences Po mercredi dernier, et encore, aujourd’hui, celle du campus de Saint Étienne. C’est pourquoi, aussi, des réunions publiques sont parfois interdites,

Le rétablissement d’un climat serein et, surtout, le respect des principes de la République font partie des priorités que l’État a fixées à l’administration provisoire de Sciences Po. Ce sera un point important du contrat

À chaque fois, à chaque nouvel incident, on s’indigne, on s’émeut, on condamne, on promet même des sanctions. Et, en définitive, on se félicite du retour au calme. Je vous le dis : il faut que cela cesse. je vous le demande : qu’y a t il derrière la ligne rouge ? Moi, je vous le dis : en France, on ne dialogue pas avec les terroristes ni avec leurs soutiens ; on n’ouvre pas de débat avec ceux qui veulent déconstruire nos valeurs et nos principes, avec ceux qui promeuvent l’islamo gauchisme dans nos universités, ceux qui agitent le feu et la haine dans une résurgence de l’antisionisme, ce faux nez de l’antisémitisme. Il est temps d’identifier, de condamner et de bannir les véritables ennemis de la République. La parole

Les avances et les hypothèses brutales concernant la réduction des dépenses publiques se succèdent et font saigner d’inquiétude les oreilles de nos concitoyens, des élus locaux et des hommes et des femmes qui travaillent dans la fonction publique territoriale. Pourtant, la part des dépenses des collectivités françaises est nettement inférieure à la moyenne européenne. Pourtant, nos collectivités sont exemplaires, qu’il s’agisse de la dette, de l’investissement ou des services publics. Les nuages s’accumulent à la suite de vos décisions vos décisions : la quasi disparition de l’autonomie financière et fiscale ; la compression des dépenses de fonctionnement de 0,5 point, en dessous de l’inflation ; les transferts de charges nets ; les transferts de compétences et de recettes qui ne sont que partiellement couverts, à l’image de la

collectivités, préconise le télétravail, alors que nous défendons le lien humain, qui est absolument indispensable, encourage les fermetures d’école, alors que nous défendons les services publics, et, enfin, évoque la sobriété foncière, ignorant le coût de la densification et du renouvellement urbains. Monsieur le ministre, ma question est simple : quel sort le Gouvernement entend il réserver aux collectivités territoriales ? La parole

Monsieur le ministre, vous n’avez pas pris position sur le rapport de l’inspection générale des finances : j’en déduis que vous en partagez les orientations. Nous le disons et redisons à chaque séance : les élus locaux ont besoin de visibilité pour leurs finances et pour leur budget. C’est un impératif démocratique, au niveau local comme au niveau national.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour le groupe Les Républicains. Ma question s’adressait à M. le Premier ministre. « Travailler moins pour gagner plus » : voilà ce qui semble être le nouveau slogan du Gouvernement. Depuis lundi dernier, les cheminots, qui, déjà, partent à la retraite plus tôt que les autres salariés, savent qu’ils pourront toucher pendant quinze mois 75 % de leur salaire sans travailler. Les contrôleurs aériens, quant à eux, ont obtenu des jours supplémentaires de récupération placés sur un compte épargne temps, utilisable pour partir en préretraite avant 59 ans. Le chantage a donc payé.

qui a relevé l’âge de départ à la retraite à 64 ans, ces accords conclus entre syndicats et directions auront un coût qui, comme toujours, sera supporté par les clients et les contribuables. Monsieur le Premier ministre, alors que vous demandez aux Français de travailler plus et plus longtemps pour redresser nos comptes publics, comment pouvez vous accepter que des entreprises publiques, sous votre contrôle, prennent le chemin inverse ?

en conduisant les propriétaires à effectuer des travaux de rénovation énergétique inadaptés, voire à délaisser ou à démolir leur bien. En France, environ 33 % des logements relèvent de ce bâti ancien, qui, une fois qualifié de « passoire thermique », risque de tomber en déshérence et de sortir du parc locatif. À l’heure où notre pays connaît une grave crise du logement, peut on vraiment se le permettre ? C’est un autre sujet.

Même si l’on sent une volonté d’avancer sur ce sujet, certains enjeux fondamentaux restent en suspens : la création d’un DPE spécifique, qui ne concernerait que le bâti patrimonial et qui reconnaîtrait enfin ses qualités ; l’évolution de la liste des travaux éligibles aux aides, primes et dispositifs fiscaux, afin que les afin que les travaux respectueux du bâti ancien soient mieux et davantage pris en compte ; enfin, un meilleur accompagnement technique et financier des collectivités territoriales dans l’identification de leur bâti patrimonial, notamment de celui qui ne bénéficie pour l’instant d’aucune forme de protection. J’aurais souhaité demander à Mme la ministre ce qu’elle pense pouvoir mettre en œuvre pour que le petit patrimoine, celui qui a traversé les siècles résisté à tous les aléas, celui qui raconte tant de notre histoire et de nos savoir faire, ne fasse pas les frais de la transition énergétique.

Vous avez raison, le DPE ne prend pas suffisamment en compte les matériaux anciens dans les modalités de calcul de la performance énergétique. C’est la raison pour laquelle la ministre de la culture travaille en étroite collaboration avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour un meilleur accompagnement et une meilleure formation des diagnostiqueurs. Aujourd’hui, le bâti patrimonial fait partie de l’examen théorique de sélection. Ce n’était pas le cas auparavant. Le temps de formation initiale a plus que doublé et comporte une session spécifique pour le bâti ancien. En dépit des études montrant que les matériaux sont vertueux, avec notamment une meilleure inertie, ainsi qu’un confort d’été et une résistance thermique souvent sous estimés, les immeubles construits avant 1948 restent souvent mal pris en compte par le DPE. La ministre de la culture entend bien évidemment, comme vous l’avez souligné,

Merci